La séance est ouverte.

site internet. La parole est à M. Hervé Marseille, pour le groupe Union Centriste. Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, le Président de la République et la Chancelière allemande ont formulé lundi une proposition ambitieuse, qui répond à l'impérieux besoin de relance économique de notre continent

alors que le fossé entre le nord et le sud de l'Europe s'était dangereusement creusé et que nous avons fortement déploré la réaction tardive de l'Europe au début de la crise. Encore faut-il que cette proposition soit approuvée par les Vingt-Sept. Mais la volonté est là des deux côtés du Rhin, et c'est déjà beaucoup puisque nous léguerons à nos enfants une dette d'une ampleur inégalée, cet argent doit être utile à un horizon qui dépasse de loin celui de la sortie immédiate de la crise. De même, l'effort consenti par les États membres impose d'utiliser ces fonds dans une perspective de long terme qui serve les intérêts de notre continent. Monsieur le Premier ministre, nous savons aussi que, pour convaincre certains de nos partenaires instruits par des décennies de mauvaises habitudes et de facilités, il nous faudra leur donner des assurances solides- ils nous connaissent trop bien ... Dès lors, comment pouvez-vous garantir que cet argent magique sera utilisé en vue de porter des investissements stratégiques nécessaires pour recouvrer notre souveraineté, préserver notre environnement et notre santé ?

République voilà deux jours. Elle fait suite à l'épidémie de Covid-19, à la crise sanitaire que l'Europe a connue à des titres divers, et à la crise économique et sociale qui s'annonce, conséquence directe à la fois du confinement lié à la crise sanitaire et à l'arrêt de la production et de la consommation que nous avons constaté dans un très grand nombre de pays d'Europe et du monde. Je vous rappelle ce ce chiffre édifiant : près de la moitié de l'humanité confinée- on entrevoit bien les conséquences économiques et sociales qui vont en découler ... Est-ce que l'Europe a été à la hauteur de la crise ? Beaucoup de nos concitoyens en France, beaucoup de nos amis en Espagne, en Italie et ailleurs diront volontiers que tel n'a pas été le cas. Auront-ils raison ? Autrement dit, les réponses de l'Union européenne, au-delà de la perception de nos concitoyens, auront-elles été à la hauteur ? Probablement pourrons-nous affirmer avec un peu de recul que l'Union européenne n'a pas rien fait et qu'elle a été utile dans la crise. Mais est-ce que, véritablement, elle a été à la hauteur de cette crise ? Je ne le crois pas, monsieur le président Marseille. Comme toujours, lorsque nous nous retrouvons dans une situation de crise, de difficultés, il faut soit le constater, vivre avec et, le cas échéant, le déplorer, soit trouver des solutions pour y remédier. Bien souvent, lorsque la crise européenne est là, c'est dans la capacité de la France et de l'Allemagne

C'est très précisément ce qui s'est passé ou, plus exactement, ce qui est en train de se passer, puisque la France et l'Allemagne se sont mises d'accord pour un plan très ambitieux, sans précédent, visant à permettre le financement d'une relance à hauteur de 500 milliards d'euros, grâce à la nouvelle capacité de la Commission à créer de la dette de façon à alimenter le marché, l'investissement, la relance.

pilier, la création d'un instrument qui permette une solidarité entre les États européens, et donc entre les citoyens européens, un fonds de relance doté, je l'ai dit, de 500 milliards d'euros de dettes émises par la Commission. Ce fonds fonctionnerait, pour l'essentiel, dans les premières années du prochain cadre pluriannuel de financement que l'Union discute et viendrait lui-même en complément des 500 milliards d'euros de prêts agréés par l'Eurogroupe. l'Eurogroupe. Les sommes en jeu sont vertigineuses et, au fond, assez peu concevables : 1 000 milliards d'euros pour financer la relance et la solidarité, auxquels s'ajouteront les dispositifs nationaux, qui se conjugueront ou compléteront le dispositif européen.

et nous renforçons nos capacités de long terme et notre capacité, à long terme, à répondre aux questionnements de nos concitoyens. Enfin, le quatrième pilier va, là encore, dans le sens de ce que vous indiquez, me semble-t-il, à savoir le renforcement de la souveraineté européenne. En effet, cette crise sanitaire cette crise sanitaire a montré que, si nous voulions maîtriser notre destin, il fallait que, dans l'espace européen, un certain nombre de productions soient localisées, qu'un certain nombre de marchés sensibles soient maîtrisés et qu'un certain nombre de dispositifs sans lesquels nous ne pouvons pas faire face aux difficultés soient assurés. C'est sur le principe de cette souveraineté européenne que la France et l'Allemagne viennent de s'entendre ; c'était le sens des annonces du Président et de la Chancelière. Il n'y a pas eu de précédent à ce type d'annonces. Pourquoi ? Parce que, et je le dis avec beaucoup de plaisir et de satisfaction, l'Allemagne a bougé

est là et que chacun peut la mesurer. Je n'exclus pas, mais sans doute ce point-là sera-t-il sujet de longues discussions, que l'Allemagne ait bougé parce que la France elle-même a bougé. Je n'exclus pas que l'Allemagne ait bougé parce qu'elle a vu que la France, en s'attaquant à des réformes de structure qui avaient parfois été évoquées, mais pas réalisées, voulait effectivement préparer l'avenir sérieusement. Je ne l'exclus tellement pas que c'est la seule raison que j'identifie pour pouvoir faire fonctionner de nouveau ce moteur franco-allemand dont nous savons tous qu'il est indispensable au redémarrage de l'Europe, non pas simplement à sa souveraineté, mais à son existence. C'est donc une excellente nouvelle qui ressort de cette annonce conjointe par le Président de la République et la Chancelière : une excellente nouvelle, pour nous, Français, pour les Allemands aussi, j'en suis certain, et pour les Européens dans leur ensemble. La vie est ainsi faite que ces excellentes nouvelles, qui ne sont pas encore traduites dans les faits- vous avez raison, car il va falloir convaincre, mais j'ai observé, vous aussi sans doute, monsieur le président Marseille, que la Banque la Banque centrale européenne et la Commission européenne s'étaient félicitées de cette annonce et de cette initiative. C'est un excellent début ! Il va évidemment falloir parler et convaincre l'ensemble de nos partenaires. C'est normal, mais reconnaissons ensemble que, lorsque la France et l'Allemagne s'accordent, lorsque, ensemble, elles avancent, en général elles entraînent. C'est une excellente nouvelle

La crise sanitaire nous a contraints, comme beaucoup d'autres pays, à organiser un confinement de la population. Il a en grande part paralysé l'économie française pendant huit semaines. Les trésoreries et l'activité de nombre d'entreprises ont été mises à mal. Et nous ne sommes qu'au début d'une crise économique Dès l'apparition de cette pandémie, le Gouvernement a mis en place des moyens exceptionnels pour faire face au choc économique, afin d'aider les entreprises et les salariés à affronter les difficultés provoquées par la Covid-19 chômage partiel, développement du télétravail, fonds de soutien, fiches métiers, guides de branches pour garantir la santé au travail, protocole de déconfinement, etc. Parce qu'il faut faire repartir l'économie et parce qu'il faut garantir la santé des salariés, l'État se doit de s'inscrire dans cette continuité et d'accentuer la reprise. C'est pourquoi votre ministère confie au réseau Anact-Aract (Association un dispositif d'appui gratuit destiné aux entreprises de moins de 250 salariés, avec un enjeu : concilier santé au travail et performance. Depuis hier, ces TPE-PME peuvent, grâce au dispositif « Objectif reprise bénéficier de préconisations gratuites qui reposent sur trois modalités d'appui : sensibilisation, conseil et accompagnement. Madame la ministre, pouvez-vous nous détailler ces modalités d'appui, nous garantir que ce dispositif est simple d'accès et prévoit des solutions accessibles à tous, en particulier aux plus petits, afin de répondre de manière optimale à leurs attentes en cette période de reprise qui suscite de très grandes inquiétudes ? La parole

arrêter ou ralentir très fortement le moteur de l'économie pour sauver des vies. Nous avons eu raison de le faire. Désormais, avec le déconfinement, nous sommes capables de continuer à sauver des vies, tout en faisant repartir l'activité économique et en protégeant pleinement les salariés. C'est pour cela, vous l'avez cité, que nous avons mis en place le protocole de déconfinement, à savoir 64 guides métiers élaborés avec les professions, avec les partenaires sociaux, par le ministère du travail, en liaison avec le ministère de la santé, et qui sécurisent

représentant 28 % de l'ensemble des consultations médicales, contre 0,1 % quelques semaines plus tôt. L'épidémie de Covid-19 a sans aucun doute provoqué un regain d'intérêt pour les solutions de télémédecine, apparues comme un outil indispensable dans un contexte de contagiosité, de confinement et d'isolement. Le succès récent de la télémédecine s'explique également par la mobilisation massive et rapide de moyens pour répondre aux besoins les plus urgents. Vous avez ainsi levé, pour le remboursement des téléconsultations Covid-19, l'obligation de passer par son médecin traitant et d'avoir eu une consultation en présentiel dans les douze mois précédents.

Face aux avancées rapides de ces dernières semaines, il n'est pas pensable de revenir à la situation d'avant Covid-19, tant les attentes sont fortes de la part des professionnels de santé, des élus et des patients. Des freins restent encore à lever. Je pense notamment au déploiement du très haut débit, dont les zones blanches coïncident souvent avec les zones sous-dotées. Je pense aussi aux nombreux trous dans la raquette s'agissant des motifs de remboursement et de la nomenclature des actes. Je pense bien sûr au financement des innovations grâce à l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2018,

est passé au cours du mois de mars de 10 000 à 500 000 par semaine, soit de 1 % à 11 % de l'ensemble des consultations. En 2018, quand ces sujets ont commencé à se présenter, les prévisions pour l'année 2020 étaient effectivement d'un million de consultations pour toute l'année un million, c'est le nombre de téléconsultations qui ont été réalisées la semaine dernière ! Outre la télémédecine, il y a aussi le télésoin. Or, vous l'avez évoqué, nous avons assoupli un certain nombre de dispositions pendant cette crise, notamment pour rendre le télésoin plus facile pour les infirmiers, les kinés, les orthophonistes, les orthoptistes, les ergothérapeutes, les psychomotriciens ou encore les pharmaciens. Dès avant la crise, le numérique est apparu comme un axe de transformation majeure pour ce gouvernement, puisque, depuis le début du quinquennat, vous le savez, nous avons engagé un certain nombre de chantiers ambitieux autour de la gouvernance de ce secteur nouveau- c'est un point important -de l'espace numérique en santé pour les usagers. Je citerai notamment le dossier médical partagé, le déploiement d'un bouquet de services numériques pour les professionnels de santé, qui en est un peu le pendant, et, bien sûr, le Health Data Hub que nous avons lancé pour tout ce qui a trait à l'innovation et à la recherche en santé. Nous serons vigilants au cours des semaines et des mois à venir pour examiner ce qui pourra être pérennisé et ce qui devra être amélioré. Je n'ai pas de doute que toutes ces réflexions-là nourriront les échanges qui s'ouvrent dans le cadre du Ségur de la santé, lancé

dans le numérique en santé aussi, il y aura un avant et un après Covid-19 ; soyez-en convaincue

Mais force est de constater que nous ne serons pas tous égaux devant cette souffrance. Des plans de suppressions d'emplois sont déjà envisagés et tombent comme des couperets : Airbus, Alinéa, Airbnb, la SNCF, TUI France ; la liste n'est malheureusement pas exhaustive. Ce sont ainsi des milliers de salariés qui vont subir un véritable tsunami social. Comment accepter qu'Air France et Renault aient bénéficié de milliards de prêts et envisagent aujourd'hui des licenciements ? Pourquoi avez-vous refusé, comme nous l'avions proposé, de conditionner ces aides à des critères sociaux et environnementaux ?

Pis, certains groupes opportunistes profitent de la crise pour orchestrer un chantage odieux auprès de leurs salariés, comme chez Derichebourg : soit les salariés reviennent sur tous leurs conquis sociaux, soit c'est un vaste plan de licenciement de 750 personnes ! Et que dire de ces groupes dont les restructurations étaient prévues avant la pandémie et qui en profitent pour les justifier, comme chez General Electric ? Il faut agir par la loi, car, sinon, après le chômage partiel, ce sera le chômage de masse, d'autant que, depuis 2017, les plans sociaux peuvent être activés au seul motif économique, qu'il soit passager ou artificiel. Plutôt que de casser le code du travail, nous vous proposons d'interdire les licenciements comme en Espagne, et, en même temps, de préparer un vaste plan de relance qui s'appuie sur la relocalisation de notre industrie, la nationalisation des entreprises stratégiques et la nécessaire transition écologique. Madame la ministre, « Les Jours heureux » ne se convoquent pas dans les discours, ils se mettent en oeuvre au prix d'une ambition politique de haut vol pour être à la hauteur de la crise que nous traversons.

l'emploi. C'est pour cela que nous avons déployé un système d'activité partielle, de chômage partiel, massif, inédit, jamais connu en France, le plus protecteur d'Europe et qui, pour ces trois mois, a protégé

je souhaite tout d'abord saluer ici le dévouement et le travail des élus locaux, qui ont fait face à ce contexte inédit de crise épidémique. Comme l'ensemble du pays, les collectivités et leurs régies sont aux prises avec des difficultés financières sans précédent. Le manque de recettes se chiffre dès à présent en dizaines de milliards d'euros. Il est du devoir de l'État de ne pas abandonner les collectivités, pour lesquelles la baisse de recettes, notamment fiscales, risque d'engloutir leur épargne, qui ne représente pas moins de 46 milliards Sans soutien important de la part de l'État, le redémarrage économique que tout le monde souhaite ici ne pourra s'effectuer dans de bonnes conditions. Vous le savez, par la commande publique, les collectivités représentent 70 % de l'investissement public dans les territoires. Ces acteurs locaux sont un maillon essentiel pour sortir du marasme actuel. Or la confiance nécessaire à l'action publique ne sera pas au rendez-vous s'ils constatent que, pour les deux à trois années à venir, leurs capacités de financement sont sérieusement diminuées. À crédits constants, les collectivités ne pourront pas jouer leur rôle moteur, alors que de nouvelles équipes municipales portent de nombreux projets de développement économique. Votre intervention récente au Sénat devant la commission des finances semblait indiquer que vous étiez consciente de la situation critique que nous traversons. Alors, concrètement, madame la ministre, quelles garanties immédiates pouvez-vous donner aux élus locaux qui veulent relancer l'économie de leurs territoires par l'investissement ? La parole est à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

des avances sur les douzièmes de dotation globale de fonctionnement, mais aussi de fiscalité, afin de soutenir la trésorerie des collectivités qui en auraient besoin.

elles seront étudiées par le Gouvernement dans la perspective d'un nouveau projet de loi de finances rectificative à venir- prochainement -, qui comportera des mesures en faveur des collectivités territoriales. territoriales. Notre action ne s'arrête bien sûr pas à ce budget rectificatif : le projet de loi de finances pour 2021 sera également un moment essentiel, puisque les pertes de recettes engendrées par la crise se feront sentir à court, à moyen et à long terme de façon différée, si je puis dire. Le débat budgétaire pour 2021 comprendra aussi une réflexion sur l'investissement dans nos territoires. Aujourd'hui comme demain,

pendant le confinement. Dans du 14 avril, un journaliste observe que chaque juridiction a construit son propre plan en fonction de ses particularités en matière de contentieux et d'organisation. C'est le maintien de l'activité pénale d'urgence et le contentieux des libertés qui prime. La justice civile, c'est une autre affaire D'après cet article, aucune chambre civile ne se réunit pour délibérer, malgré la procédure sans audience prévue par une ordonnance du 25 mars. Ayant longtemps été avocat moi-même, j'ai tenté de vérifier les informations contenues dans cet article en effectuant un très rapide et modeste tour de France des juridictions, afin de ne pas m'arrêter sur le ou les tribunaux qui auraient dysfonctionné.

Ils ont déploré que le système informatique utilisé par les avocats avec les greffes, RPVA, ne soit pas accessible par les magistrats travaillant à leur domicile sur leur portable. Ils ont considéré que la sécurité sanitaire mettait en conflit plusieurs vérités concurrentes : la santé des personnes- des magistrats, des avocats, des greffiers, mais aussi des justiciables, le service des justiciables en droit de la famille ; la santé économique des cabinets d'avocats, du fait du problème posé entre autres par l'aide juridictionnelle. Ils ont relevé que des dysfonctionnements nombreux, mais pas généralisés, liés au droit de retrait de certains magistrats, ont rendu impossible l'organisation d'audiences et occasionné des retards de jugement. de jugement. Une mission d'information serait nécessaire, une après-midi d'enquête ne suffit pas. Ma question est donc nourrie par des réponses variées, plutôt constructives : quelles leçons entendez-vous tirer de cette période, madame la garde des sceaux, afin de permettre un fonctionnement de la justice mieux adapté aux crises ? La parole est à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

La parole est à M. Michel Raison, pour le groupe Les Républicains. Les soignants n'ont pas attendu l'épidémie pour démontrer leurs compétences. Les Français qui ont eu à connaître l'hôpital avant la crise sanitaire tenaient déjà en haute estime le personnel soignant, car ils mesuraient déjà le dévouement des aides-soignants, des infirmiers, des médecins, des brancardiers, des agents de nettoyage. Depuis des mois, unanimement, ces personnels appelaient à l'aide et dénonçaient leurs conditions de travail. Ne commettons pas une nouvelle erreur de diagnostic : le mal est profond, le mal est ancien. La réponse ne doit être ni contextuelle ni provisoire, ce qui serait pire. Prescrire médailles et participation à un défilé guerrier est dans le meilleur des cas une blague de mauvais goût, dans le pire, une pique incendiaire. Le Président de la République a annoncé un plan pour l'hôpital, dont on ignore tout pour le moment. Nous souhaitons tous en connaître les contours et son articulation avec l'ensemble des acteurs de santé. Nous nous méfions des discours de théâtre. Ce plan sera-t-il pensé de façon locale, articulé autour des territoires et des professionnels de santé, qui sont au plus près des malades, mais aussi des dysfonctionnements organisationnels ? Êtes-vous prêts à engager une véritable décentralisation de la décision

de ceux qui nous soignent. C'est en partant de leur expérience, notamment pendant cette crise, que nous devons bâtir le plan pour l'hôpital que vous avez évoqué. Chacun devra y être associé

a parfois confirmé des choses que nous savions. Elle a aussi parfois bousculé nos certitudes. Elle a permis de l'inventivité, de la créativité, de nouvelles pratiques. C'est tout cela que nous voulons, monsieur le sénateur, faire remonter des territoires pour bâtir l'hôpital de demain. Les Français aspirent à une protection sociale qui soit forte,

plus rapidement. Il n'y aura pas de sujet tabou, par exemple sur l'articulation entre le public et le privé. Les agences régionales de santé, que vous avez évoquées et que vous connaissez bien,

par la fermeture ou la transformation à court ou moyen terme de plusieurs sites, dont celui de Flins-sur-Seine principalement. Monsieur le Premier ministre, l'État est un actionnaire important du groupe Renault, il ne méconnaît donc en rien ses intentions. Le plan de soutien et de relance du secteur automobile annoncé par Bruno Le Maire serait fondé sur un modèle « plus durable ». Le site de Flins-sur-Seine, qui s'appuie sur un écosystème puissant de sous-traitants locaux, sur la proximité d'un centre de recherche au véhicule autonome et propre, est le site de production emblématique de ZOE, au coeur d'un territoire d'industrie que vous avez récemment mis en place. Il est donc le site idéal pour servir de point de départ à une stratégie de transformation vers plus de durabilité. Il ne saurait en être autrement. D'ailleurs, vous allez probablement octroyer dans les jours qui viennent un prêt garanti de l'État de 5 milliards d'euros à Renault

la sécurisation de sa trésorerie et de ses capacités d'investissement devient un enjeu majeur. L'État, vous l'avez dit, est au rendez-vous pour l'accompagner.

Il est toujours mieux en de telles circonstances de franchir plus vite encore les étapes que l'on prévoyait de franchir plutôt que d'essayer de défendre le plus longtemps possible une position qui serait en vérité intenable.

Nous ne supportons plus la désindustrialisation continue de notre territoire et nous sommes prêts à investir auprès de l'État et de Renault pour assurer cette transformation dans notre département. La parole est à M. Bernard Jomier, pour le groupe socialiste et républicain. Monsieur Monsieur le secrétaire d'État, le 26 février dernier, j'interrogeais Olivier Véran dans cet hémicycle sur les moyens attribués aux hôpitaux et aux professionnels de ville pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

N'en restez pas aux mesures parcellaires et homéopathiques de votre prédécesseur. La réponse doit nous conduire à rétribuer nos personnels soignants comme un pays européen qui place la santé publique au premier rang de ses priorités. Quand annoncerez-vous des décisions en la matière ? Un second tempo impose de repenser l'organisation de notre système de soins, de revoir la place, les missions et l'organisation de l'hôpital et de redéfinir en particulier ses moyens en fonction de ses missions, et non l'inverse. Le Président de la République a, à demi-mot, semblé admettre les carences de la loi de 2019, laquelle n'a pas su défaire les méfaits du concept d'« hôpital-entreprise ». C'est un premier pas. Il faut aussi redéfinir l'articulation avec les acteurs de ville et médico-sociaux, écartés pendant près de deux mois de la gestion de l'épidémie, par une décision prise au sommet, alors qu'ils ont bien souvent démontré leur sens de l'adaptation au plus près du terrain, leurs capacités à aller vers les populations et les territoires les plus touchés, fondement de toute réponse efficace à une épidémie. Sur ces chantiers, un nouveau catalogue de mesures, un nouveau projet de loi parachuté d'en haut avec des experts serait une nouvelle erreur. À cet égard, les déclarations d'Olivier Véran il y a quelques heures ne nous rassurent pas. Il faut maintenant organiser des états généraux impliquant l'ensemble des acteurs, dont les Français bien sûr.

Je sais que vous suivez avec attention tous ces sujets depuis longtemps. Je sais aussi que vous avez passé plusieurs semaines durant la crise à l'hôpital de Melun. Je ne

est claire : nous allons augmenter les rémunérations des personnels soignants ; cela a été dit à plusieurs reprises par le Président de la République, par le Premier ministre, par le ministre de la santé. Nous allons proposer un plan d'investissement ambitieux. Vous savez qu'il était déjà question d'une reprise importante de la dette des hôpitaux, mais d'autres voies peuvent être explorées en complément. Nous allons engager une transformation profonde de tout ce qui ne tire pas l'hôpital et la santé de nos concitoyens vers le haut. Notre seule contrainte, monsieur le sénateur,

Dans un communiqué publié le 11 mai, M. le ministre de la santé a cependant réaffirmé sa volonté d'accorder une prime à cette

des aides à domicile sur tout le territoire puisque le financement de cette prime dépendra de l'état budgétaire de chaque département. Il serait donc injuste que ces salariés pâtissent de la gouvernance dont ils dépendent. La crise sanitaire a démontré leur dévouement, leur écoute ; ils forment un maillon essentiel dans la chaîne des soins. Par leur mobilisation, ils ont contribué à ce que l'hôpital ne soit pas submergé. Ils étaient présents, travailleurs de l'ombre, d'aucuns diraient « invisibles de la République ». La réalité est là : ils souffrent d'une faible rémunération, de l'ordre de 900 euros nets par mois, qui n'est pas en adéquation avec l'effort qu'ils Monsieur le secrétaire d'État, ma question est simple : allez-vous attribuer à cette profession, dans des conditions de justice et d'égalité territoriale, une prime financée par l'État et équivalente à celle que vous comptez verser aux personnels des Ehpad ? La parole

Il faudra que nous en terminions enfin avec ces silos entre la médecine de ville, l'hôpital, le secteur médico-social et le social, et que nous puissions à l'avenir avoir des réponses plus uniformes. heures. Mes chers collègues, par courrier en date du 19 mai, M. le Premier ministre m'a informé que le Gouvernement fera, en application de l'article 50-1 de la Constitution, une déclaration, suivie d'un débat et d'un vote, relative aux innovations numériques la lutte contre l'épidémie de Covid-19, mercredi 27 mai, le soir. En conséquence, la suite de l'examen du projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne est reportée au jeudi 28 mai, à l'issue de l'ordre de jour réservé au groupe socialiste et républicain et, éventuellement, le soir. Acte est donné de cette demande. Après concertation avec les présidents de groupe et le Gouvernement, nous pourrions prévoir, à la suite de la déclaration du Gouvernement, un temps attribué aux groupes politiques réparti de la manière suivante : sept minutes pour les groupes Les Républicains, socialiste et républicain et Union Centriste, minutes pour les autres groupes et trois minutes pour les sénateurs n'appartenant à aucun groupe. Après la réponse du Gouvernement s'ouvrirait une séquence de onze questions-réponses, à raison de trois questions pour le groupe Les Républicains, deux questions pour les groupes socialiste et républicain et Union Centriste et une question pour les autres groupes. Il n'y a pas d'observation ? ... Il en est ainsi décidé.